la commission des affaires sociales demande au Sénat, en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête, pour une durée de six mois, afin de mener une mission d'information sur l'adéquation du passe vaccinal à l'évolution de l'épidémie de covid-19.

citoyen et écologiste. Monsieur le ministre, le Président de la République a lancé, aujourd'hui, devant le Parlement européen, la présidence française du Conseil de l'Union européenne (PFUE). Les défis à relever sont nombreux. Mais l'échec social est au coeur des crises qui déchirent l'Union, laquelle a été longtemps réduite à un vaste champ d'application du principe de mise en concurrence, où le progrès social est sacrifié. Aujourd'hui, face aux pandémies, au dérèglement climatique, aux inégalités, tout esprit lucide admet que l'Europe doit changer de trajectoire. Le temps est venu de passer du logiciel du « tout pour le marché, la concurrence et la finance » à celui du « tout pour la solidarité, l'humain et la planète

La France proposera-t-elle de sortir les dépenses publiques et de recherche consacrées à la santé des critères soumis à l'examen du semestre européen ?

Monsieur le sénateur Laurent, si vous me le permettez, je crois que c'est plutôt au parti communiste de changer de logiciel

Quel est le continent qui a le mieux protégé ses entreprises et évité des centaines de milliers de faillites pendant la crise la plus grave que nous ayons eu à connaître depuis 1929 ? C'est le continent européen. Quel est le continent qui, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, a décidé de lever de la dette en commun pour la première fois de son histoire, afin de financer des mesures de protection et de relance économique face à la crise ? C'est le continent européen. Quel est le seul continent au monde actuellement une réflexion sur un salaire minimum commun ? C'est le continent européen. Quel est le seul continent au monde qui est en train de se doter de normes de protection environnementale en réfléchissant, sous présidence française,

Alors, regardez l'Europe telle qu'elle est, monsieur le sénateur, et voyez à quel point elle a changé. Apportez votre soutien à cette Europe solidaire et efficace que nous sommes en train de construire avec le Président de la République La parole est à M. François Patriat, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

pays. Entre 2017 et 2021, la France a maintenu ou créé 140 000 emplois autour de projets qui font de l'attractivité de la France un élément indispensable aujourd'hui.

continuer la politique économique et sociale que nous conduisons au service de la France et les Français ! La parole est à M. Thierry Cozic, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Tout le monde l'aura compris : la seule réponse que vous êtes en mesure d'apporter face à la flambée des prix de l'énergie relève au mieux de l'improvisation, au pire du cynisme électoral. Vous faites peser sur EDF l'entière responsabilité de la soutenabilité financière des mesures gouvernementales de campagne. Après avoir tardivement compris que votre chèque énergie de 100 euros n'aurait que peu d'effets face à la hausse des prix, vous vous êtes aventurés dans d'autres dispositifs. Votre décision pourrait coûter 8 milliards d'euros à EDF, alors que l'urgence est de financer le renouvellement et l'entretien du parc productif. Force est de constater que le marché de l'énergie en France est devenu le royaume de la financiarisation : le parc de production d'électricité n'a jamais été réellement agrandi et la production d'énergies renouvelables stagne toujours. trente-cinq sont des fournisseurs virtuels, qui ne produisent pas un kilowatt et spéculent à partir des approvisionnements garantis par EDF, le tout en empochant la différence, et que l'on retrouve domiciliés dans des paradis fiscaux. Monsieur le ministre, quand allez-vous mettre en oeuvre les mesures nécessaires afin d'arrêter de subventionner une concurrence factice, qui se développe au mépris de l'intérêt général et qui ne contribue qu'à l'enrichissement privé ?

choisir. Notre choix, nous l'avons déjà fait : protéger les Français contre l'augmentation massive des prix de l'électricité et protéger nos entreprises contre une augmentation insupportable de leurs coûts de production.

affaire à des responsables politiques qui tiennent leurs promesses ! Le Premier ministre avait promis que les tarifs de l'électricité n'augmenteraient pas de plus de 4 % pour les consommateurs français. Promesse tenue ! Ce sera le cas et cela nous change de la politique du passé Monsieur le ministre, votre réponse ne me convainc pas. Je vous parle des problèmes systémiques et structurants d'EDF, et vous n'apportez qu'une réponse conjoncturelle. Le marché de l'énergie est devenu en France un gigantesque far west financier, qui ne sert que ses intérêts ! Où est l'intérêt public dans tout cela ? Cette spéculation est une lame de fond, qui grève le pouvoir d'achat de nos concitoyens et place EDF dans une situation intenable pour les années à venir. Avec cette opération, vous détruisez notre fleuron industriel. Comme le dit l'adage, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Avec cette mesure, monsieur le ministre, vous venez d'« enrager » EDF, et c'est bien regrettable

Cette situation touche plus particulièrement les secteurs de l'hôtellerie-restauration, du BTP, de l'industrie, du commerce, de la santé et du grand âge, des transports et de la logistique.

pour lesquels nous manquons de candidats, et des emplois peu qualifiés, pour lesquels un vivier de main-d'oeuvre existe, mais dont l'attractivité fait défaut. Ces deux situations nécessitent des mesures différenciées mieux adapter l'offre de formation au marché du travail et améliorer les conditions d'emploi. Cet automne, le Gouvernement a d'ailleurs lancé un plan fondé sur ces deux principes pour réduire les tensions en termes Mais, d'après l'avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE), les politiques en la matière doivent cibler un spectre bien plus large. Au-delà des mesures pour renforcer l'attractivité des métiers, telles que les hausses de salaire, l'existence de freins périphériques à l'emploi. C'est pourquoi il souligne l'importance d'une politique globale touchant au logement social, aux solutions d'accueil des jeunes enfants ou encore à la couverture du territoire en transports collectifs. Aussi, madame la ministre, allez-vous adapter votre plan de lutte contre les difficultés de recrutement et associer les collectivités locales à une politique à la fois plus globale et plus adaptée à chaque territoire ? La parole

en matière de recrutement peuvent être source de difficultés pour les entreprises, mais elles constituent aussi une bonne nouvelle, car elles sont le signe que la reprise est robuste. Il nous faut donc accompagner cette reprise en répondant aux besoins de main-d'oeuvre des entreprises, qui constituent autant d'opportunités pour les jeunes et les demandeurs d'emploi. Depuis le début du quinquennat, nous investissons comme jamais dans la formation : je pense notamment au plan d'investissement dans les compétences à hauteur de 15 milliards d'euros. Plus récemment,

Comme vous l'avez signalé, il convient également de renforcer l'attractivité des métiers en tension. C'est le sens des discussions que j'ai engagées avec certaines branches pour les inciter à revaloriser leur minima conventionnels et à améliorer leurs conditions de travail. La branche des hôtels, cafés, restaurants a ainsi réussi à proposer une hausse moyenne des salaires de plus de 16 %. Comme le souligne le CESE dans son avis, il nous faut aussi lever l'ensemble des freins périphériques au retour à l'emploi. C'est avant tout à l'échelon local que des réponses peuvent être trouvées en partenariat avec les collectivités. Nous avons donc demandé à chaque sous-préfet d'identifier, avec les acteurs locaux, les solutions qui peuvent être proposées aux demandeurs d'emploi, en tenant compte des spécificités des territoires. Enfin, il nous faut nous assurer que les demandeurs d'emploi à qui ces formations sont proposées s'en saisissent effectivement et répondent aux offres d'emploi. C'est tout le sens du contrôle de la recherche d'emploi, qui a conduit à une radiation de près de 18 % des demandeurs d'emploi contrôlés au cours du mois de décembre. Monsieur le sénateur, l'ensemble de ces actions commencent à porter leurs fruits. Ces derniers mois, les embauches ont atteint un niveau inégalé depuis près de vingt ans.

et Territoires. Madame la ministre, « on ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants ». Ces propos du Président de la République ont choqué les étudiants et le personnel de l'université. Si le but est de faire baisser la précarité étudiante en rendant l'université moins accessible aux plus précaires, c'est inacceptable ! Cette vision de l'université s'inscrit dans la continuité d'un mandat plus que décevant les dépenses par étudiant ont ainsi continué de baisser ; le bilan de Parcoursup est plus que mitigé ; l'université souffre d'un sous-financement chronique et les conditions d'encadrement des étudiants ne cessent de se dégrader

Pour nous, l'éducation est au coeur d'une société de l'intelligence, de la solidarité, de l'épanouissement et de l'émancipation. Tout comme l'hôpital, elle doit rester gratuite

ce que nous avons fait depuis 2017 ! Il propose également de demander aux universités de mieux travailler à l'insertion professionnelle, à la formation continue, à la formation tout au long de la vie, et de le faire évidemment avec les futurs employeurs des étudiants. Voilà le projet que nous défendons depuis cinq ans. Madame la sénatrice,

Comme eux, nous voulons une réforme des bourses, des investissements massifs dans l'université publique et la mise en place d'une allocation autonomie. Vos propos ne sont pas une réponse à la hauteur des attentes des étudiants et des universités. La parole

le 13 janvier dernier, le Gouvernement demandait à EDF d'augmenter de 20 % le volume de l'électricité issue de la filière nucléaire vendue à prix réduit à ses concurrents dans le cadre de l'accès ce afin de contenir à 4 % la hausse des tarifs. Cette décision, dont le coût est évalué à ce jour à 8 milliards d'euros, dessine de sombres perspectives pour un fleuron national déjà lourdement fragilisé.

gouvernementales pour sauvegarder le pouvoir d'achat des Français sont louables, elles suscitent nombre d'interrogations et d'inquiétudes, notamment dans cet hémicycle. Elles vont aussi largement profiter aux concurrents d'EDF, sans certitude que cela se répercute sur leurs clients. Monsieur le ministre, EDF doit faire face à beaucoup trop d'injonctions contradictoires : fermeture de Fessenheim, renouvellement du parc nucléaire, grand carénage et, aujourd'hui, mise à contribution pour contrer la hausse du coût de l'énergie. du coût de l'énergie. Cette équation insoluble met en danger l'entreprise et compromet gravement son avenir. À l'heure où tout le monde parle de souveraineté énergétique et où la France prend la présidence du Conseil de l'Union européenne, quelles perspectives entendez-vous tracer pour EDF, qui concourt depuis 1946 à la stratégie énergétique de la France ? Comptez-vous donner à EDF les moyens de ses ambitions ?

Maintenant, nous voulons ouvrir des perspectives de long terme. La première a été rappelée par le Président de la République : nous entendons faire d'EDF un des leaders mondiaux de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Il est temps ! Le Président de la République, le Premier ministre,

Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, la transition énergétique ne se fera pas sans EDF. Enfin, nous l'espérons- après ce que nous venons d'entendre, nous commençons effectivement à douter ... Il ne se passe pas un mois sans que votre gouvernement prenne des décisions fragilisant EDF.

la Pentecôte ! Mais plus encore, c'est sur l'intégrité même du groupe EDF qu'il y a le plus d'inconnues, puisque nous ne savons toujours pas ce que vous voulez faire de notre opérateur national- et je ne parle pas des incertitudes sur les barrages. Ma question est simple, monsieur le Premier ministre, au-delà des belles paroles que nous venons d'entendre, avez-vous décidé de sacrifier EDF ?

que la seule solution était d'augmenter le plafond de l'Arenh, afin que, dans une telle configuration, le dispositif de prix aidé fonctionne de manière efficace.

Les autorités maliennes n'en sont plus à une provocation près. Elles continuent de nier la présence des mercenaires russes dans le pays, allant même jusqu'à remettre en cause le survol de leur territoire par les appareils de transport logistique intervenant au profit de l'opération Barkhane, et ce malgré un accord de coopération datant de 2013.

À la fin de l'année dernière, Paris laissait entendre que le report des élections maliennes prévues le mois prochain, mais surtout l'arrivée du groupe Wagner seraient « inacceptables ». Force est de constater que nous avons été mis devant le fait accompli. Avec le redimensionnement de la force Barkhane, se posera également la question de la mission des Nations unies pour la stabilisation du Mali et le déploiement de la force Takuba. Neuf ans après le début de l'opération militaire au Sahel, le Mali remet en cause la présence française sur son sol. Plus le temps passe, plus les États contributeurs- européens, en particulier -vont se poser des questions. Pouvons-nous durablement envisager une présence sur un territoire où nous ne sommes plus les bienvenus ? Dans ces conditions, et à la suite de la réunion à Brest des ministres des affaires étrangères des Vingt-Sept, quelle position la France et Bruxelles entendent-elles adopter ?

la présence avérée du groupe Wagner au Mali est un symptôme de la fuite en avant dans laquelle la junte s'est engagée. Comme la Cédéao l'a relevé, la junte tente de prendre en otage le peuple malien pour les cinq prochaines années. C'est absolument inacceptable ! Wagner est présent au Mali, non pas pour lutter contre le terrorisme- il ne l'a jamais fait en Afrique -, mais pour assurer le maintien au pouvoir de la junte. Dans ce contexte, les chefs d'État de la Cédéao ont pris à l'unanimité des décisions fortes et courageuses fermeture des frontières et de l'espace aérien malien, arrêt des transactions commerciales et financières, gel de l'assistance financière de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Il revient maintenant à la junte de poser des actes pour se conformer aux engagements pris, au risque de s'enfermer dans un isolement régional et international. L'Union européenne appuie très résolument, et de manière unanime, ces décisions fortes de ses partenaires africains. C'est le sens des discussions que le ministre Jean-Yves Le Drian a eues avec ses homologues européens lors du Gymnich de Brest. L'Union européenne va prendre des sanctions individuelles contre les responsables de la junte malienne, qui entravent le processus de transition. Je rappelle qu'elle a d'ores et déjà pris ses responsabilités, en adoptant des sanctions au mois de décembre contre le groupe Wagner, ses cadres dirigeants et ses entités.

pour la réplique. Monsieur le ministre, la présence française au Mali se complique de jour en jour. Nous ne sommes pas parvenus à nous opposer à l'arrivée des mercenaires russes. Il y a désormais urgence à prendre des décisions fermes contre la junte, qui refuse de céder le pouvoir, comme elle s'y était engagée, dans le cadre d'une transition démocratique. La parole est à M. Pierre Charon, pour le groupe Les Républicains. Madame la ministre, Madame la ministre, au-delà du saccage de Paris dû au manque de coordination des chantiers, des travaux et de la voirie défoncée, la situation parisienne en matière de circulation et de stationnement n'est plus acceptable En voulant redéfinir les compétences en matière de circulation et de stationnement entre la mairie et le préfet de police, la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain a en réalité introduit de la complexité dans un dispositif devenu complètement illisible. Avant cette loi, qui aura bientôt cinq ans, la rédaction des articles concernés avait le mérite de ne prévoir qu'un seul régime. Qu'il s'agisse de motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens, le préfet de police était compétent en matière de circulation et de stationnement sur les voies parisiennes. La nouvelle répartition des compétences entre la maire et le préfet n'a pas réglé les difficultés à Paris, bien au contraire. Que constate-t-on ? En dépit d'une baisse de trafic automobile, les bouchons ont considérablement augmenté. Paris serait devenue en 2019 l'une des villes au monde connaissant le plus d'embouteillages. Dès 2017, le préfet de police avait pourtant prévenu des difficultés d'intervention des véhicules de secours, mais aussi de police, notamment dans le cadre de l'interdiction de toute circulation automobile sur la rue de Rivoli. Concernant le périphérique parisien, qui draine chaque jour plus de 250 000 voitures, il a fallu que le préfet intervienne pour éviter que celui-ci ne passe immédiatement à une À deux ans et demi des jeux Olympiques, des mesures législatives et réglementaires doivent être prises si l'on ne veut pas que l'événement se transforme en un énorme bouchon parisien. Il est urgent, madame la ministre, que l'État reprenne la main au plus tôt sur ces questions de circulation et de stationnement à Paris, afin de faire en sorte que Mme Hidalgo arrête d'« emmerder » les Franciliens et les Parisiens.

ne dispose plus que d'une compétence d'exception aux abords des sites dits sensibles de la capitale. Comme vous, j'observe les grandes difficultés- pour ne pas dire son incapacité -de l'actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo, à réussir à se saisir de cette compétence. Toutefois, aux termes de la convention de coordination de la police municipale de la Ville de Paris et des forces de sécurité de l'État du 13 octobre 2021, la police municipale assure, à titre principal,

Prenez le métro ! ... et soulèvent des difficultés pour les services de secours et d'intervention. Nous sommes donc, tout comme vous, monsieur le sénateur, très préoccupés par la situation, qui est du ressort de la mairie de Paris, en application du choix du législateur de 2017 de transférer l'essentiel de la compétence de circulation et de stationnement au maire de Paris.

que la présence de la société Wagner n'était pas compatible avec la manière dont la France concevait la lutte contre le terrorisme au Mali. Nous sommes d'accord. Depuis le 23 décembre, des doutes s'effacent quant à l'implication de Wagner sur le théâtre malien. La presse rapporte les premiers accrochages de ses miliciens au début de l'année 2022, près de Bandiagara. Les faits sont là, les hommes de Wagner se déploient au Mali : ils ont été repérés à Ségou. Le silence du gouvernement malien ne pourra pas masquer longtemps le concert barbare de ces mercenaires, dans un conflit dont la complexité ne saurait être résolue par l'usage d'une milice à la solde de l'argent. Seule l'instabilité en sortira gagnante et les conséquences seront graves pour les populations maliennes, d'autant que la junte ne prévoit plus d'élections et décide désormais de confisquer le pouvoir. La ligne rouge a été transgressée, c'est un fait !

Carlotti, pour la réplique. C'est Jean-Yves Le Drian, lui-même, qui a défini la ligne rouge, monsieur le ministre. Maintenant que nous y sommes, il donne l'impression de ne pas avoir de solution. C'est cette improvisation qui nous inquiète ! Nous sommes à un niveau de tension rarement atteint, ayant contraint le Président de la République à annuler son déplacement à Bamako

À l'heure du bilan, la « révolution » est bien là, mais ce n'est pas celle que les Français espéraient ! Partout dans notre pays, en ville comme à la campagne, ce sont, non pas des émeutes comme aurait pu s'en émouvoir Louis XVI, mais bel et bien des révolutions orchestrées par des voyous. ces cinq années, aucun territoire n'a été épargné- c'est une élue de Lot-et-Garonne qui le dit. Chaque jour, c'est un torrent de faits divers, de délits, de crimes, qui viennent nourrir l'actualité. Oui, la grande leçon de ce quinquennat, c'est bien la faillite d'Emmanuel Macron sur le plan régalien : fort avec les faibles, faible avec les forts, le Président de la République a totalement déserté je souhaite poser au Gouvernement sont simples. Que regrettez-vous de ne pas avoir fait pendant ce mandat en matière de sécurité ? Êtes-vous vraiment fiers de cette société fracturée, abîmée, que vous allez laisser aux Français ?

Cette grande loi permettra de consolider les avancées du pays en matière de sécurité et les propositions des parlementaires seront évidemment les bienvenues pour la compléter. La parole tout va très bien, madame la marquise ! Pourtant, la réalité est la suivante : 1 agression toutes les 44 secondes ; 38 % d'augmentation des agressions sexuelles depuis 2017 ; trois fois plus d'agressions et de menaces contre les élus depuis 2019

Union Centriste. Ma question s'adresse à M. le ministre des solidarités et de la santé, que mon groupe interrogeait déjà en juillet 2020 sur le projet de plateforme des données de santé des Français, le Health Data Hub,

choix imposé par son collègue Cédric O, sans appel d'offres spécifique, au prétexte incroyable qu'il n'existerait aucune entreprise française ou européenne capable ! J'alertais sur les risques pour nos libertés publiques d'un tel choix, la crise sanitaire ayant, en plus, mis une loupe sur ce sujet hypersensible des données de santé.

pleinement mobilisées pour accompagner les projets de recherche, notamment sur sa plateforme technologique. En accord avec le ministère, le Health Data Hub a retiré provisoirement sa demande d'autorisation pour héberger la base principale du système national des données de santé. Cette décision est prise dans un contexte où la CNIL a commencé à instruire l'arrêté définissant la composition de ces bases de données, sensibles par essence. Cette instruction, une fois finalisée, consolidera l'ensemble du dispositif de mise à disposition des données, comme prévu par le décret de juin 2021. Nous souhaitons assurer notre souveraineté sur les données de santé des Français et nous poursuivrons ce déploiement à compter du moment où ces conditions de confiance et de sécurité seront réunies. Entre-temps, nous mobilisons tous les leviers disponibles pour avancer. Le ministère a demandé à l'assurance maladie, en lien avec cette plateforme, d'élaborer un plan d'action pour accélérer la fourniture des données liées au système national concerné. Les premiers résultats sont déjà là, avec une centaine de projets pour 2021, témoignant à la fois de la très forte demande et de l'utilisation croissante des données. Notre objectif, qui sera précisé au cours du mois de janvier, est de doubler le volume de données mises à disposition pour les projets de recherche, afin de concilier les attentes des porteurs de projets. Le Health Data Hub se met donc bien en place ; il n'est pas à l'arrêt et porte ses premiers fruits. Mais ces avancées sont réalisées dans un cadre légal sécurisé et renforcé par les avis de la CNIL, avec le soutien constant du Gouvernement. Nous ne faisons pas de pari sur les données de santé des Français. Nous voulons des résultats tangibles pour notre recherche, dans un cadre sécurisé et de confiance. Madame la ministre, vous ne m'avez pas répondu sur la question financière, qui est très importante. Quel est le coût de cette plateforme, censée permettre à terme des économies ? Nous venons d'apprendre que l'assurance maladie refusait de verser sa quote-part de 11,5 millions d'euros

La parole est à Mme Valérie Boyer, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le ministre, ma question porte sur les « menaces de mort » du président autocrate de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, à l'encontre de notre candidate Valérie Pécresse lors de son déplacement en Arménie et en Artsakh. Je veux saluer sa démarche sincère et courageuse, cohérente avec ses engagements. Valérie Pécresse, Michel Barnier et Bruno Retailleau se sont rendus à plusieurs reprises au chevet des chrétiens d'Orient, des Yézidis et des Kurdes en Irak, au Kurdistan, témoignant un soutien que nombre d'entre nous ont aussi C'est le Parlement, avec Gérard Larcher, Bruno Retailleau, l'ensemble des groupes du Sénat, qui a été l'honneur de la diplomatie française, le 25 novembre 2020, en faisant voter une résolution et en nous rendant dès le mois d'avril 2021 en Artsakh. Alors que la France préside le Conseil de l'Union européenne, le silence du Gouvernement est d'autant plus condamnable et inquiétant. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une réponse en catimini du chef de l'État, qui nous rappelle la loi en vigueur dans cette dictature, ne la condamne même pas et ne soutient pas ses élus. Pourquoi ne pas exiger des excuses solennelles de l'Azerbaïdjan ?

Jean-Yves Le Drian l'a hier très clairement rappelé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale : ces propos sont inacceptables. Cette position du gouvernement français a d'ailleurs été rappelée à l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en France. Pour autant, je veux vous le dire, nous n'avons pas attendu le déplacement de Mme Pécresse pour agir en solidarité avec le peuple arménien et pour faire en sorte que la crise dans cette région du monde s'apaise.

Ces efforts se poursuivent aujourd'hui, en lien avec l'Europe, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Je vous rappelle que le Président de la République a réuni à Bruxelles, le 15 décembre dernier, le premier ministre Pachinian et le président Aliyev pour justement rechercher des solutions à ce conflit. madame la sénatrice, sans polémique, sans essayer d'instrumentaliser quoi que ce soit dans une visée électorale, qui est notre responsabilité. La parole monsieur le ministre, l'ambassadeur azerbaïdjanais nie toujours ces menaces et nous nargue en considérant que Valérie Pécresse n'a pas respecté la loi azerbaïdjanaise sur un territoire qui ne lui appartient même pas, en diffusant des et des photos truquées. Mais qui a violé les lois en bombardant civils et églises, en utilisant des armes interdites, en ne rendant pas les prisonniers de guerre ? Qui qualifie nos alliés arméniens de « chiens » ? Qui envoie des mercenaires djihadistes ? Qui menace la paix en attaquant ce territoire souverain qu'est l'Arménie ? Valérie Pécresse s'est rendue en Artsakh, car elle croit en la dignité des peuples, elle croit aux nations souveraines, qui doivent maîtriser leurs décisions et protéger leur peuple et leur civilisation. Valérie Pécresse préfère la sobriété de l'action, la fidélité à ses engagements plutôt que l'agitation, la communication et les compromissions. Comme de nombreux parlementaires qui sont rendus en Artsakh, comme Jaurès au Parlement en 1896, Valérie Pécresse a voulu témoigner en femme d'État : « Quoi, devant tout ce sang versé, devant ces abominations et ces sauvageries, devant cette violation de la parole de la France et du droit humain, pas un cri n'est sorti de vos bouches, pas une parole n'est sortie de vos consciences, et vous avez assisté, muets et, par conséquent, complices, à l'extermination complète. » Monsieur le ministre, en tant que membres du groupe de Minsk, nous ne pouvons plus nous réfugier derrière cette neutralité ; être neutre, c'est choisir son camp, et jamais nous ne pourrons choisir celui de la dictature et de l'abjection.

et Républicain. En France, chaque année, 100 000 jeunes quittent le système scolaire sans diplôme ni qualification.

2022 a été proclamée Année européenne de la jeunesse ; c'est aussi le trente-cinquième anniversaire d'Erasmus. Or, dans le programme de la présidence française, une seule présidence, une seule proposition concrète : le service civique européen. Mais je m'étonne et je me demande d'ailleurs si vous le savez : le service volontaire européen existe depuis vingt ans déjà et a été transformé en 2018 en corps européen de solidarité. Alors, quel est le sens de cette annonce ? Demain, devant l'agence Erasmus+ France seront présentées les propositions issues des consultations « jeunes » dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe : visiblement, ils aspirent à du concret

La Commission a publié le 14 octobre dernier une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur une Année européenne de la jeunesse pour 2022. Cette initiative est destinée à mieux accompagner les jeunes dans la sortie de la crise sanitaire et à les aider à surmonter son impact négatif. Cette décision fixe quatre objectifs, que je vais rappeler et que nous aurons à coeur de mettre en oeuvre.

entendons encourager tous les jeunes, en particulier ceux qui sont issus des milieux défavorisés, à devenir des citoyens actifs et engagés ainsi que des acteurs du changement. Je pense là bien sûr à l'engagement civique. promouvoir les possibilités offertes par les politiques publiques, au niveau européen, national, régional et local, afin de soutenir leur développement personnel, social et professionnel dans un monde vert, numérique et, surtout, inclusif. Enfin, il s'agit d'intégrer la politique de jeunesse dans tous les domaines pertinents de la politique de l'Union, afin d'encourager la prise en compte du point de vue des jeunes dans l'élaboration des politiques publiques à tous les niveaux. Il s'agit de la clause d'impact jeunesse, que nous appliquons déjà. Madame la sénatrice, à l'occasion de cette présidence, la France sera aux côtés des institutions européennes, des États membres et de l'ensemble des parties prenantes pour piloter, à l'échelle européenne, durant ces six mois, quelques sujets d'intérêt pour la jeunesse européenne et, bien sûr, pour les mettre à l'ordre du jour du Conseil. Je pense évidemment au soutien à la mobilité des jeunes dans un autre pays de l'Union européenne afin qu'elle soit plus inclusive, et ce en lien avec les annonces du Président de la République française sur le service civique européen. Vous l'avez dit, nous fêtons d'ailleurs aujourd'hui les trente-cinq ans d'Erasmus. Il faut conclure ! Je pense également au mentorat, sujet sur lequel le Gouvernement travaille et qui pourrait être porté à l'échelle européenne. La parole

Je vous parlais du service volontaire européen ; vous me répondez en vous référant à une annonce du gouvernement français sur le service civique, qui existe déjà. Il s'agit là donc d'un effet d'annonce, d'un gadget. Une politique de la jeunesse ne se mène pas à coups d'annonces ou de gadgets. Elle suppose une politique de fond, qui s'inscrit dans la durée. Elle suppose surtout d'accompagner les acteurs associatifs et de leur permettre d'être encore plus performants pour l'implication dans les programmes européens, ce qu'ils essayent de faire depuis trente ans. C'est un enjeu de taille, mais c'est un enjeu qui vaut le coup. Ce matin, le Président disait qu'il fallait faire de l'Europe une puissance démocratique, culturelle et d'éducation. On ne peut pas faire l'impasse sur la jeunesse pour aboutir à ce résultat.

Madame la ministre, il y a un an, le 27 janvier 2021, je vous interpellais en séance- comme aujourd'hui -sur l'inquiétude des communes de station de nos massifs montagneux quant à leurs difficultés budgétaires et de trésorerie. Des réponses ont été apportées par les lois de finances pour 2021 et de finances rectificatives de juillet 2020 et de juillet 2021, mais rien ne leur a été versé, ou si peu, et sans commune mesure par rapport aux pertes subies et aux dépenses nouvelles de gestion de la crise sanitaire. Si des compensations ont été apportées aux professionnels de la montagne, ce dont chacun se félicite, les communes n'ont pas été compensées des pertes de recettes de taxes professionnelle et touristique-

Ces exemples, madame la ministre, vous les connaissez puisque vous avez vérifié auprès des trésoreries la véracité des plaintes des maires de communes de montagne. Pour la seule année 2021, une perte de 500 000 euros pour Saint-Lary-Soulan, dans les Hautes-Pyrénées de plus de 300 000 euros pour Isola, dans les Alpes-Maritimes ; de 1 million d'euros pour Valloire ; de 5 millions d'euros pour Bourg-Saint-Maurice, en Savoie. La commune Les Belleville, sur 6 millions d'euros de pertes, a perçu un acompte de 100 000 euros en novembre 2021, la base de 30 % de la somme perçue en 2020, ce qui représente, vous le voyez, une somme dérisoire au regard des pertes réelles. Admettez que cette situation n'est pas tenable. Ces communes, qui se demandent comment équilibrer leur budget de fonctionnement surdimensionné pour la population touristique,

effectivement, les finances des communes montagnardes ont été lourdement mises à contribution, dès 2020, et de manière très marquée en 2021, avec la fermeture des remontées mécaniques l'hiver dernier. Par conséquent, plusieurs mesures de compensation ont été prises.

fixé à partir de janvier. Olivier Dussopt et moi-même avons adressé des consignes en ce sens au préfet de la Savoie, et certains dossiers complexes comme celui des Belleville sont en voie de règlement. Le Premier ministre l'a écrit à l'Association nationale des maires des stations de montagne représentants relaient ce message auprès des élus. Deuxièmement, je rappelle que nous avons indemnisé de nombreux services et équipements publics gérés en régie-

a indemnisé les pertes d'activité des exploitations de remontées mécaniques, même si celles-ci sont gérées en régie publique, dans les mêmes conditions que nous l'avons fait pour le privé. Voilà, en quelques mots, madame la sénatrice, des éléments factuels qui montrent bien que nous sommes aux côtés des stations de montagne.

Courageux face à la maladie, tout comme sa famille, ce petit garçon est depuis quelques jours au coeur de l'actualité. Alors que le processus médical touchait à sa fin et qu'on espérait une issue heureuse, le petit Joseph a fait une rechute. Les parents, désespérés, lancent un appel aux donneurs de moelle osseuse les réseaux sociaux. Sans ce don, Joseph ne survivra pas. Cet appel a largement été repris par les médias. Monsieur le secrétaire d'État, à votre tour, allez-vous le relayer avec les moyens de la puissance publique ? Au-delà du drame vécu par Joseph et sa famille, cette question pose le problème de la rareté des donneurs volontaires inscrits au registre international dédié. La pénurie est endémique : l'Agence de la biomédecine recherche en permanence de nouveaux donneurs. Certains freins administratifs sont incompréhensibles : alors que l'on peut donner sa moelle osseuse jusqu'à 60 ans, on ne peut s'inscrire sur ce registre qu'entre 18 et 35 ans. Pourquoi pas plus tard, alors que c'est le cas dans d'autres pays ? Mais le principal obstacle au développement du fichier des donneurs est le manque d'information. Les gens ignorent l'étendue des besoins et de nombreuses idées reçues perdurent. À titre d'exemple, pour être inscrit dans le fichier des donneurs, il suffit de procéder à un prélèvement salivaire ou sanguin. Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement va-t-il prendre les mesures nécessaires pour, enfin, faciliter le don de moelle osseuse et lancer une campagne d'information pour développer le fichier des donneurs ?

je suis évidemment sensible, comme chacun d'entre vous ici, aux situations individuelles dramatiques et à la situation du petit Joseph, que vous avez rappelée et que vous me donnez d'ores et déjà l'occasion, comme vous l'avez fait, de mettre en lumière. Il est

entre deux individus pris au hasard. C'est la raison pour laquelle l'Agence de la biomédecine gère le registre France greffe de moelle, qui recense 320 000 donneurs et qui est connecté à ceux de 73 autres pays. Cela permet donc d'avoir accès à 40 millions de donneurs potentiels.

plus rapide pour les patients, avec une efficacité non pas garantie, mais en tout cas plus assurée. Par ailleurs sont visés les hommes, car les cellules souches de leur moelle osseuse sont dépourvues des anticorps que développent les femmes durant leur grossesse.

La liberté d'expression est un principe fondamental de notre République » : voilà ce que déclarait Gérald Darmanin en novembre 2020. Ministre de l'intérieur, vous êtes le garant de nos libertés, qui sont protégées par les forces de l'ordre, que vous dirigez. Vous, monsieur Darmanin, vous n'étiez pas à Ibiza ; vous avez donc dû voir passer l'information selon laquelle plusieurs interventions de parlementaires contre le passe vaccinal ont été censurées par YouTube ou Facebook. S'il n'y a plus de délit de blasphème en France, les GAFA (Google, Apple, Facebook, Bastien Lachaud, député LFI, mon collègue de l'Assemblée nationale Nicolas Meizonnet et moi-même en avons été victimes. Alors, qu'ils s'en prennent au président des États-Unis, il y a deux ans, c'était déjà limite. Mais s'en prendre à moi, monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, vous conviendrez quand même que, là, ça va trop loin À l'aube d'une campagne présidentielle cruciale pour l'avenir du pays, les Français ont besoin d'être assurés que leur principale source d'information, les réseaux sociaux, demeurera libre. Nos personnes ne sont pas sacrées, mais notre liberté d'expression, elle, l'est, en particulier dans les hémicycles du Parlement, le coeur même de notre démocratie. Pendant des mois, on a essayé de nous faire peur avec une prétendue « ingérence russe », qui allait renverser les urnes du monde libre. La réalité, c'est que la seule ingérence étrangère, de plus en plus totalitaire, vient non pas du Kremlin, mais de la Silicon Valley, de quelques milliardaires en jeans-baskets reçus comme des chefs d'État à l'Élysée, qui veulent influer sur les élections grâce à leur entreprise planétaire. Vous n'avez donné aucune garantie depuis cinq ans à ce sujet, alors même que vous avez fait passer une loi contre les fausses informations. À ce titre, monsieur le ministre de l'intérieur, vous en avez vous-même propagé une ce dimanche, faisant croire que des manifestants contre le passe vaccinal défilaient le bras tendu, alors qu'ils étaient en train de réaliser un, c'est-à-dire de taper dans leurs mains comme cela se fait dans tous les stades de France. Alors, monsieur le ministre, ma question est double : après cet épisode navrant, qui démontre que vous avez décidé vous aussi d'« emmerder » les non-vaccinés jusqu'au bout, jusqu'au bout du, que comptez-vous faire pour protéger la liberté d'expression et ne craignez-vous pas d'être condamné, à votre tour, pour propagation de fausses informations ?

D'abord, je veux vous dire que la liberté d'expression sur les réseaux sociaux comme la liberté d'expression dans la vie n'est pas infinie ; elle est encadrée par la loi. Par exemple, diffuser de fausses informations ou inciter des gens à mettre leur vie en danger ne relève pas de la liberté d'expression.

ne relève pas de la liberté d'expression, monsieur le sénateur. Oui, nous sommes attachés à la liberté d'expression, à la liberté d'expression des parlementaires, et, dans cet hémicycle, bien évidemment, elle est pleine et entière. C'est pourquoi nous pouvons y avoir cet échange, comme en dehors de celui-ci. Mais la liberté d'expression n'est pas sans limite. C'est pourquoi nous avons fait adopter des lois pour faire en sorte, par exemple, qu'on ne puisse pas, au nom de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, y diffuser l'adresse personnelle d'un professeur ou d'un policier en menaçant leur vie,

La séance est reprise. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein des commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale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 L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à renforcer le droit à l'avortement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

Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure- chère Laurence Rossignol -, mesdames, messieurs les sénateurs, nous reprenons aujourd'hui les débats sur ce sujet nous reprenons aujourd'hui les débats sur ce sujet sensible et éminemment important qu'est le renforcement du droit à l'avortement, même si- et j'anticipe -nos discussions seront probablement abrégées par l'adoption d'une motion présentée par votre commission des affaires sociales.

Mais nous fallait-il encore des exemples pour nous rappeler que le droit à l'avortement est loin d'être garanti pour toutes les femmes et que ce droit, chèrement acquis il y a tout juste quarante-sept ans, doit toujours être affirmé, protégé, renforcé En outre, la crise sanitaire que nous traversons nous impose une plus grande vigilance encore pour que les droits sexuels et reproductifs soient garantis et que le droit inaliénable à l'avortement soit pleinement effectif. Le retour devant votre Haute Assemblée de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement est l'occasion pour le Gouvernement de réaffirmer son engagement plein et entier à défendre sans relâche le droit des femmes à avorter en toute sécurité, dans le respect de leur choix éclairé par un accès à des informations fiables, objectives et au plus près de leur lieu de vie.

sans possibilité d'exercer son droit. À cet égard, je souhaite vous indiquer où en sont les engagements qui ont été pris devant la représentation nationale. Tout d'abord, les délais pour réaliser une IVG médicamenteuse en ville seront prolongés jusqu'à sept semaines de grossesse et le parcours pourra être réalisé en fonction du choix et de l'état de santé des femmes par téléconsultation. Le ministre des solidarités et de la santé s'était engagé à faire entrer ces mesures dérogatoires prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dans le droit commun. Le processus est en cours. La Haute Autorité de santé, saisie en septembre 2020, a actualisé ses recommandations en avril 2021 sur le parcours d'IVG médicamenteuse, en confirmant la prolongation des délais et le recours à la téléconsultation. Le décret d'application est prêt et est examiné en ce moment même par le Conseil d'État ; il devrait donc pouvoir être publié très rapidement. Les IVG instrumentales en centre de santé peuvent désormais être mises en oeuvre, le décret en précisant les conditions ayant été publié en avril dernier. Le cadre de l'expérimentation pour la réalisation des IVG instrumentales par les sages-femmes en établissement de santé a fait l'objet d'une concertation et a été finalisé avec les professionnels, médecins et sages-femmes. Le décret d'application a été publié le 31 décembre 2021. les sages-femmes, la formation et l'expérience requises, ainsi que l'organisation spécifique exigée des établissements de santé expérimentateurs. Il est accompagné d'un arrêté, qui organise l'appel national à candidatures auprès des établissements de santé volontaires. Cette démarche doit conduire à la sélection d'une cinquantaine d'équipes et au lancement des tout premiers projets d'ici au milieu de l'année Elle constitue une étape importante pour poser les bases d'une pratique, qui, sans nul doute, facilitera l'organisation des équipes hospitalières pour répondre aux demandes d'IVG et offrira aux femmes un nouvel interlocuteur dans leur parcours d'IVG. Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le tiers payant intégral obligatoire est dorénavant prévu pour toutes les femmes sur les dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire, soit 100 % des frais liés à l'IVG, dans le cadre de forfaits de prise en charge. s'ajoute la garantie du respect du secret quant à la prise en charge de ces frais pour toutes les femmes. Dans les deux assemblées, les parlementaires ont également souligné la nécessité de faire progresser l'information et l'éducation à la vie intime et affective, et globalement de promouvoir plus fortement la santé sexuelle. Le Gouvernement fait pleinement siens ces objectifs. Ainsi, la feuille de route 2021-2024 de déclinaison de la stratégie nationale de santé sexuelle, résultat d'une coconstruction avec l'ensemble des parties prenantes, a été publiée le 1 décembre dernier. nombre d'actions concrètes pour renforcer la promotion, l'information et l'éducation à la santé sexuelle. Il s'agit, par exemple, de la conception et de la diffusion d'outils de promotion de la santé sexuelle accessibles aux publics en situation de handicap

et comprend une action dédiée au renforcement de l'accès à l'IVG, car nous devons toujours conforter l'exercice effectif de ce droit en tout point du territoire. Les premières mesures concrètes ont été adoptées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Je pense à l'extension de la consultation longue « santé sexuelle » à tous les jeunes jusqu'à 25 ans, pour que la santé sexuelle cesse d'être vue comme une affaire de femmes. Je pense également à l'accès gratuit à la contraception pour les femmes jusqu'à 25 ans, pour tenir compte des vulnérabilités économiques et sociales des jeunes adultes. Enfin, je tiens à rappeler la place essentielle de la profession de sage-femme dans nos politiques de prévention et de santé des femmes, mais aussi des hommes. Qu'il me soit permis, à cet effet, de souligner les avancées de la loi Rist (loi du 26 avril

le Gouvernement est fier d'assurer aujourd'hui une reconnaissance tant attendue par les plus de 20 000 représentants de cette profession, pour renforcer comme jamais l'attractivité de ce métier et sa place dans nos politiques publiques, tout particulièrement en santé sexuelle et reproductive. Mesdames, messieurs les sénateurs, en décembre 2020, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE), que le Gouvernement avait souhaité saisir sur la question de l'allongement du délai légal, qui met en jeu le droit des femmes, leur santé, aussi bien que le rôle des professionnels et l'accès à l'IVG, a rendu son avis. seulement l'importance des mesures de protection des femmes et de prévention des grossesses non désirées, mais aussi la nécessité de renforcer l'éducation affective, à la santé sexuelle et reproductive. Le CCNE précise que, si la réalisation des IVG comporte des risques qui augmentent avec l'âge gestationnel, ces derniers sont néanmoins faibles et diffèrent peu entre douze et quatorze semaines semaines de grossesse. Enfin, en axant sa réflexion sur les principes d'autonomie, de bienfaisance, d'équité et de non-malfaisance à l'égard des femmes, le CCNE a considéré qu'il n'y avait pas d'objection éthique à allonger le délai d'accès à l'IVG de deux semaines. Toutefois, pour faire progresser concrètement le droit des femmes à disposer de leur corps, il faut résolument poursuivre l'amélioration de leur parcours, afin que les IVG dites « tardives » soient mieux prises en charge, et sans délai. C'est un droit des femmes ; c'est notre devoir, c'est notre responsabilité à tous de permettre à chacune son plein exercice, selon son choix, sa situation et son lieu de vie.

le Gouvernement défend farouchement ce droit des femmes, ce droit humain tout simplement, garanti par notre Constitution. Notre devoir est de le renforcer et d'améliorer sans cesse son effectivité. Cet engagement, le Président de la République l'a réaffirmé avec force ce matin même, devant le Parlement européen, en appelant de ses voeux la reconnaissance du droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Quant à la question posée par ce texte, elle relève pleinement de la représentation nationale : le Gouvernement s'en remettra à la délibération qui résultera des débats parlementaires et, donc, à votre sagesse.

décidé de déposer une motion tendant à opposer la question préalable. Je reviens sur le contenu du présent texte, que nous commençons tous à connaître, même s'il a un peu évolué en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. L'allongement du délai de recours à l'IVG, de quinze jours, jusqu'à la fin de la quatorzième semaine de grossesse, a été maintenu, ce qui permettrait à notre pays de s'aligner sur les délais légaux en vigueur dans d'autres États européens.

Sont également en cause des cycles irréguliers, l'absence de signes cliniques et des changements graves intervenus dans leur vie matérielle, affective ou sociale.

J'y vois une reconnaissance bienvenue et attendue de la filière maïeutique, devenue centrale dans l'accès à l'IVG. Par souci de sécurité des soins, les IVG chirurgicales ne pourront être réalisées par les sages-femmes qu'en établissement de santé. Bien entendu, elles répondront à des exigences de formation et d'expérience. Je me réjouis également de la pérennisation de l'allongement du délai de recours à l'IVG médicamenteuse en ville jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse.

de 1975, entre une Assemblée nationale majoritairement hostile à l'IVG et une ministre, Simone Veil, qui voulait la dépénaliser et la légaliser.

Simone Veil a fait comme elle a pu : elle a utilisé les arguments dont elle avait besoin pour convaincre une majorité qui ne voulait pas de sa loi. Mais nous ne sommes plus en 1975, nous sommes en 2022. Le débat est un peu différent et nous avons désormais un peu d'expérience

La loi Veil, relative à l'interruption volontaire de grossesse, a marqué un tournant salutaire pour notre pays et nous sommes les défenseurs de ce droit imprescriptible. Selon une étude publiée en septembre 2020 par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, en 2019, le taux de recours a atteint 15,6 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans dans l'Hexagone. C'était là son niveau le plus élevé depuis 1990.

ce sont les jeunes qui sont touchées. En effet, 65 % des interruptions volontaires de grossesse concernent des femmes de 19 à 25 ans. Les jeunes femmes rejettent de plus en plus la pilule et les méthodes de contraception qui ne sont pas naturelles. Elles leur préfèrent le stérilet, et dans l'idéal en cuivre, pour éviter tout traitement hormonal. On observe un véritable phénomène générationnel et un changement des jeunes femmes dans leur rapport à la contraception, qu'il nous faut comprendre et analyser. Ce phénomène dépasse le seul enjeu du délai dans lequel une interruption volontaire de grossesse est possible. Les moyens que nous mettons en oeuvre pour l'accompagnement et la prévention sont insuffisants ; les campagnes d'information ne sont pas assez ambitieuses ; et nous ne parvenons pas à toucher un public parfois distant de nos moyens de communication publics. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 étend le remboursement de la contraception de 18 à 25 ans. C'est une avancée majeure, qui doit modifier notre cadre d'analyse. Légiférer à nouveau sur ce sujet sans avoir pris le temps d'analyser les effets de cette mesure, sans disposer d'aucun bilan de son impact sur le nombre d'IVG, ou plus précisément sur le nombre de demandes d'IVG hors délai,

quatorze semaines accroît les risques, notamment d'hémorragie et d'accouchement prématuré lors des grossesses ultérieures. L'Académie nationale de médecine elle-même s'est prononcée contre l'allongement du délai de recours à l'IVG, compte tenu des risques de complications pour les femmes à court et moyen termes. À mon sens, notre travail doit se concentrer sur le droit en vigueur concernant l'accompagnement des jeunes femmes. Les huit jours qui s'écoulent entre la demande d'IVG et la réalisation sont parfois vécus comme un moment très difficile. Il faut que la prise en charge des femmes soit mieux assurée dans le délai actuel.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, Simone de Beauvoir a écrit : « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis.

Alors que le Parlement européen vient d'élire à sa tête une femme farouchement hostile à l'avortement, il me semble plus qu'indispensable de réaffirmer ce droit pour que les femmes puissent, en leur âme et conscience, mettre un terme à une grossesse non désirée dans des

Certes, de nombreuses améliorations ont été apportées ces vingt dernières années- délai de recours porté de dix à douze semaines de grossesse en 2001, gratuité en 2013, suppression du critère de « situation de détresse

sous-valorisation de l'acte, disparités territoriales du fait, notamment, d'une diminution du nombre de professionnels. En 2013 déjà, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes alertait face à la fermeture de plus de 130 établissements pratiquant l'IVG. Dans ces voient évidemment le nombre de services d'orthogénie se réduire peu à peu. Au pays de Simone Veil, les obstacles sont malheureusement toujours aussi nombreux. C'est dans cet esprit que la proposition de loi dont nous débattons cette après-midi- ou, plus précisément,

allonger le délai d'accès à l'IVG de deux semaines. À son sens, il n'y a que « peu, voire pas de différence entre douze et quatorze semaines de grossesse ». Il estime toutefois que cet allongement ne doit pas servir à pallier les défaillances de notre politique publique de santé Dans ces conditions, il est légitime de se demander si l'allongement du délai légal permettra réellement aux femmes d'accéder plus facilement à l'IVG. C'est pourquoi certains sénateurs de mon groupe se montrent assez réservés, craignant que cette mesure ne soit, en fait, une mauvaise réponse à un vrai problème. Comme l'a rappelé notre rapporteure, l'allongement du délai légal ne constitue qu'une partie de la solution ; la refonte globale du pilotage de l'activité d'IVG et plus largement de notre politique de santé sexuelle et reproductive est essentielle.

Les travaux de l'Assemblée nationale ont toutefois enrichi le présent texte, notamment en permettant aux sages-femmes de réaliser des IVG chirurgicales jusqu'à la quatorzième semaine de grossesse ; en pérennisant l'allongement du délai de recours à l'IVG médicamenteuse en ville de cinq à sept semaines ; en supprimant le délai de réflexion de deux jours ; ou encore en renforçant l'effectivité des l'effectivité des sanctions auxquelles s'exposent les professionnels de santé qui refuseraient de délivrer un moyen de contraception d'urgence. Mes chers collègues, que nous soyons pour ou contre l'allongement de deux semaines du délai légal, ce sujet méritait d'être débattu et examiné de manière très approfondie. C'est pourquoi, une fois de plus, le RDSE votera unanimement contre la motion ! La parole est à M. Stéphane Ravier.

revient au Sénat par la volonté du Gouvernement, alors que le Président de la République déclarait au mois de juillet dernier dans un journal de presse féminin : « Je mesure le traumatisme que c'est », pour une femme, « d'avorter ». Et voilà ... En effet, contrairement à ce que voudrait nous faire croire Mme Rossignol, rapporteur de la commission, l'avortement n'est pas un acte anodin. L'exécutif manie donc un sujet grave au gré de ses intérêts électoraux. La réalité, c'est que ces délais sont aussi élastiques que les convictions de ceux qui les défendent. D'ailleurs, les mêmes qui s'émeuvent de propos sur les personnes handicapées élargissent sans scrupule de grossesse (IMG) jusqu'au neuvième mois de grossesse- une véritable ignominie. Alors que le pays réel manque de médecins, de maternités, de sages-femmes et de gynécologues pour accompagner la vie à naître et les femmes enceintes, le pays légal a pour seule préoccupation de faciliter l'avortement. Le pays légal, en dissonance cognitive, autorise depuis le mois de décembre 2021 à donner un prénom à l'état civil à un enfant décédé dans le sein de sa mère tout en voulant reporter le seuil de l'avortement. En 2019, la France établissait un triste record, à 232 000 avortements. En 2020, elle en totalisait 220 000, soit l'équivalent de la population de la ville de Rennes, chaque année ! Je le dis avec beaucoup d'humilité, dans cette enceinte où le débat- je crois -est permis, parce que cette réalité touche beaucoup de femmes au plus profond de leur chair, de leur coeur et de leur âme notre rôle est de permettre d'éradiquer les causes qui poussent la jeunesse, en particulier, à la désespérance. Les lois régentent toujours plus de secteurs de la vie, mais les Français n'y trouvent pas leur bonheur. en plus ... de plus en plus d'anxiolytiques et sont les leaders européens de consommation de cannabis. Quel est le rapport ? Le progressisme n'a pas élargi les horizons : il n'a fait qu'abattre des murs porteurs. Notre rôle de législateur est de réinsuffler l'espérance aux familles françaises. Or, en 2010, 47 % des femmes qui avortaient le faisaient principalement pour raisons matérielles. Ce chiffre a forcément augmenté avec la crise sociale et économique que nous subissons.

La natalité dans notre pays a connu en 2020 son niveau le plus bas depuis 1945, mais, pour les mondialistes, même humains, il ne s'agit que d'une comptabilité. La natalité française implose ? Peu importe Elle sera remplacée par une immigration qui explose, ... C'est honteux ! ... et vive la grande famille mondialisée et déracinée ! Mes chers collègues, j'avais conclu mon discours en première lecture par : « Familles françaises, je vous aime. » Je voudrais dire ici que, même si vous ne les aimez pas, vous avez le devoir de les soutenir. Elles sont l'avenir de notre pays, elles sont la nation française. Moi, en tout cas, je peux vous garantir que, personnellement, je fais le maximum

à opposer la question préalable sur ce texte. Nous nous rappelons bien qu'ici même, il y a moins d'un an, le groupe Les Républicains du Sénat avait déjà refusé tout débat en séance sur la question pourtant fondamentale du droit à l'IVG. En instaurant l'allongement du délai de recours à l'IVG de douze à quatorze semaines de grossesse, ce texte représente une réelle avancée pour le droit des femmes. Chaque année, quelques milliers de femmes se retrouvent hors délai pour avorter. Parmi ces femmes, certaines sont forcées de poursuivre leur grossesse

a considéré qu'il n'existait « que peu, voire pas de différence de risque pour la femme avortant entre douze et quatorze semaines de grossesse » et n'a donc émis aucune objection éthique à l'allongement de ce délai. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain soutient l'initiative

à supprimer le délai de réflexion- pour le moins infantilisant, il faut le dire -de deux jours, imposé afin de confirmer une demande d'avortement ; à préciser que le pharmacien refusant la délivrance d'un contraceptif en urgence sera en méconnaissance de ses obligations professionnelles ; et à créer un répertoire recensant les professionnels et structures pratiquant l'IVG. Cet ensemble de mesures représente une avancée importante. Malheureusement, le texte présente, à son retour de l'Assemblée nationale,

Comme l'a déjà évoqué à différentes reprises Mme la rapporteure Laurence Rossignol, nous devons mettre en place une politique nationale et proactive pour notre offre de soins en orthogénie et, plus largement, en matière de santé sexuelle et reproductive. Il est en effet indispensable d'améliorer l'information dans les lycées et les collèges, et de lutter contre l'absence d'éducation à la vie sexuelle et affective. Plus d'un quart des établissements scolaires n'en dispensent pas, alors que c'est une obligation. en outre de nombreuses inégalités. Il s'agit d'abord d'inégalités territoriales. Entre 2007 et 2017, 70 centres ont fermé en France métropolitaine. Ainsi, 37 départements compteraient moins de 5 professionnels de santé libéraux pratiquant les IVG médicamenteuses. Ce manque de structures et les disparités qui existent entre les territoires restreignent de fait la liberté des femmes à recourir à la méthode d'IVG de leur choix. À ces inégalités territoriales s'ajoutent celles qui sont liées au niveau de vie des femmes. d'âge et situation conjugale comparables, les femmes dont le niveau de vie se situe dans les 10 % les moins élevés ont une probabilité supérieure de 40 % de recourir à l'IVG par rapport à celles dont le niveau de vie est classé parmi les 10 % les plus élevés. élevés. Un pilotage national est donc indispensable pour organiser l'effectivité du droit à l'IVG pour toutes les femmes de France. Ce droit fondamental à l'avortement a été rappelé ce matin même par le Président Macron au niveau européen,

Cette fois encore, le Sénat ne pourra vraisemblablement pas débattre de cette question majeure, qui touche des centaines de milliers de femmes en France chaque année, puisque la commission des affaires sociales a décidé de déposer une nouvelle motion tendant à opposer la question préalable. Nous en prenons acte. Aucune femme », comme le rappelait Simone Veil à la tribune de l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974, « ne recourt de gaieté de coeur à l'avortement. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. » Toutefois, il s'agit surtout d'un droit : un droit précieux pour l'émancipation des femmes, fruit d'un long combat, un droit qui, près d'un demi-siècle après sa déclaration, fait encore l'objet d'attaques répétées, en Europe notamment, mais pas uniquement. Je pense au leader des députés européens LR, qui a indiqué au Parlement européen que l'IVG n'était pas un droit fondamental. Depuis plus d'un an, la Pologne, dont la législation est déjà l'une des plus restrictives d'Europe, a interdit l'avortement en cas de grave malformation du foetus. Alors que des milliers de femmes polonaises défilent dans les rues depuis plus d'un an pour défendre le droit à disposer de leur corps, le Parlement européen vient par ailleurs d'élire sa nouvelle présidente, ouvertement anti-avortement. Votre groupe a voté pour elle ! Quel triste symbole pour l'Europe. Quel triste symbole pour le Parlement européen, instance démocratique de l'Union européenne qui considère que les droits fondamentaux de la personne humaine ne connaissaient pas de frontière. Victor Hugo disait : « Ce que Paris conseille, l'Europe le médite. Ce que Paris commence, l'Europe le continue. » dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, l'interruption volontaire de grossesse dans la Charte européenne des droits fondamentaux, ce qui constitue une réponse forte aux attaques dont elle fait l'objet. Chaque année, selon les sources, entre 1 000 et 4 000 femmes sont contraintes d'avorter à l'étranger en raison du dépassement du délai légal de douze semaines de grossesse.

Partant de ce constat, ce texte propose ainsi d'allonger de deux semaines les délais légaux, comme cela a déjà été fait chez nos voisins espagnols. Rappelons d'ailleurs que ces délais sont bien plus élevés chez certains de nos voisins européens, puisqu'il est fixé à dix-huit semaines en Suède, vingt-deux aux Pays-Bas et jusqu'à vingt-quatre semaines au Royaume-Uni. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a retiré du texte la suppression de la clause de conscience spécifique relative à l'IVG. Je le regrette. Je le regrette, car il existe dans notre droit une clause de conscience générale, qui m'apparaît suffisante pour permettre à un médecin de ne pas pratiquer une IVG sans avoir à donner les motifs Cette modification du texte est donc pour moi un échec, puisque j'estime que cette double clause de conscience, qui fait de l'IVG un acte à part, est source de stigmatisation pour les femmes qui font le choix d'y avoir recours. Ce texte présente toutefois des avancées, que je souhaite saluer. Je pense à l'extension des compétences des sages-femmes à la pratique d'IVG instrumentales, qui permettra de renforcer l'offre médicale sur notre territoire. Je pense également à la suppression du délai de réflexion de quarante-huit heures en cas d'entretien psychosocial et à la possibilité de sanctionner un pharmacien qui refuse la délivrance d'un contraceptif en urgence. de parole pour saluer l'action du Gouvernement et la prise en charge, depuis le 1 janvier, de la contraception pour les femmes de moins de 25 ans. Une réflexion devra avoir lieu sur les disparités qui existent en la matière, puisqu'on sait que l'achat de moyens de contraception est davantage effectué par les femmes. Pour conclure, mes chers collègues, le groupe RDPI soutient, dans sa grande majorité, cette proposition de loi. Notre objectif est commun : endiguer les freins qui rendent difficile l'accès à l'IVG et garantir à chaque femme le droit à disposer de son corps. La parole est à Mme Colette Mélot.

Le texte que nous allons examiner vise à « renforcer le droit à l'avortement ». Cette formulation est équivoque, et elle peut ainsi être entendue de deux façons. La première consiste à laisser entendre que le droit à l'avortement a été affaibli. Cela n'a jamais été le cas. Depuis 1975 et l'adoption de la loi Veil, la législation a au contraire évolué afin de faciliter l'accès à l'IVG.

La deuxième façon d'entendre le renforcement du droit à l'avortement revient à considérer qu'il est encore possible de faciliter l'accès à l'IVG et de lever certains obstacles. Cette deuxième acception repose sur l'idée que la loi est encore trop restrictive et que ces restrictions empêchent concrètement certaines femmes d'exercer leur droit.

Pourquoi légiférer et couvrir ainsi le laxisme de notre société, favoriser les égoïsmes individuels au lieu de faire revivre une morale de civisme et de rigueur ? » Cette question est grave, et nous devons l'aborder sans juger les femmes qui recourent à l'IVG. En 1975, elles étaient 300 000, chaque année, à enfreindre la loi pour mettre un terme à leur grossesse, en se mettant elles-mêmes en danger. Aujourd'hui encore, de nombreuses femmes sont contraintes de partir à l'étranger lorsqu'elles ont dépassé le délai légal, pour ne pas enfreindre la loi. Nous ne pouvons l'ignorer. Sans entrer dans la bataille des chiffres- car il ne s'agit jamais que d'estimations -, nous pouvons nous accorder sur le fait qu'elles sont quelques milliers à le faire chaque année. Ce sont évidemment des milliers de trop. Personne ne peut le nier. ce chiffre doit être mis en perspective avec le nombre des avortements pratiqués tous les ans en France, autour de 230 000. Cela représente plus d'une grossesse sur quatre. Soyons-en conscients. Je le dis avec toute ma conviction : l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. » Ces mots ne sont pas les miens ; ce sont encore ceux de Simone Veil. Ce que disent les chiffres que j'ai cités, c'est que les Françaises recourent en grand nombre à l'avortement. C'est leur droit, et nous ne devons pas les juger. Il s'agit néanmoins d'un fait indéniable. C'est pourquoi je ne suis pas sûre qu'il soit nécessaire de renforcer ce droit en augmentant le délai légal- d'autant que le rallongement du délai pose problème sur le plan médical. Entre douze et quatorze semaines de grossesse, le foetus commence à se former et l'organogénèse s'accélère. La pratique de l'IVG est plus compliquée, plus risquée aussi, par la dilatation du col et l'éventualité de complications hémorragiques. La solution n'est certainement pas de contraindre les médecins qui, au regard de leur conscience professionnelle, ne veulent pas pratiquer l'acte. Ce serait même dangereux. En tout cas, il n'est pas responsable de laisser croire que l'allongement du délai d'accès à l'IVG à quatorze semaines est sans conséquence. Il vaut mieux simplifier l'accès à l'IVG avant la douzième semaine. Je crois, pour ma part, que la solution réside pour l'heure dans la prévention et l'accompagnement des femmes qui vivent une situation de détresse psychologique. Comme le disait Simone Veil, l'avortement est toujours un drame.

Parmi les mesures envisagées figure notamment l'allongement du délai légal d'interruption volontaire de grossesse de douze à quatorze semaines. Dès lors, je m'interroge : en quoi cet allongement de délai permet-il de renforcer le droit à l'avortement ? ? La question se pose de la nature des freins qui conduisent des femmes à recourir tardivement à l'avortement, au-delà du délai de douze semaines autorisé par notre législation, et qui obligeraient même certaines d'entre elles à se rendre démarche qui s'inscrirait dans la même logique que celle qui prévalait avant la loi Veil de 1975. Notre législation serait-elle si rétrograde qu'elle ne permettrait pas de répondre aux attentes légitimes des femmes, et ce en dépit des différents textes adoptés pour améliorer les conditions d'exercice de ce droit ? S'interroger sur les raisons de ces IVG tardives, qui justifieraient le passage de douze à quatorze semaines- c'est-à-dire de quatorze à seize semaines d'aménorrhée -me semble un préalable indispensable pour se positionner sur ces délicates questions. Parmi les raisons invoquées figurent la défiance des femmes, notamment des plus jeunes, à l'égard des contraceptifs hormonaux, un déficit d'information sur les méthodes contraceptives, la précarité financière et sociale, un accès déséquilibré aux professionnels pratiquant les IVG en fonction des territoires, la crise sanitaire, des diagnostics tardifs de grossesse, ainsi que des changements notables dans la situation matérielle, sociale ou affective des patientes. Il est à relever qu'en 1975, déjà, Simone Veil, dans son intervention à l'Assemblée nationale, faisait état des raisons sociales, économiques ou psychologiques des femmes ayant recours aux avortements clandestins. En dépit de l'allongement du délai intervenu en 2001, les IVG tardives reposent sur les mêmes causes qu'en 1975. C'est là une vraie question, qui doit nous interpeller fortement. Toutes ces motivations relèvent de conditions socioéconomiques défavorables et démontrent la nécessité d'adapter et de promouvoir des politiques publiques susceptibles d'apporter des réponses à ces problèmes, qui concernent évidemment l'IVG mais vont bien au-delà

En revanche, allonger le délai d'accès à l'IVG de deux semaines soulève de véritables questions spécifiques pour les femmes et pour les praticiens. Vous me permettrez de reprendre les propos du professeur Israël Nisand, que l'on ne saurait suspecter d'être un anti-IVG, puisqu'il est à l'origine de l'allongement du délai de dix Pour lui- et je partage pleinement son point de vue -, plus une IVG est tardive, plus elle est dangereuse physiquement et psychologiquement pour la patiente. Le col de l'utérus peut être dilaté davantage, induisant un risque de perforation et d'infection postopératoire, d'autant qu'il s'agit non plus d'une IVG médicamenteuse ni même d'une IVG instrumentale par aspiration, mais bien d'une IVG instrumentale chirurgicale. Quant au foetus, il mesure déjà douze centimètres, sa tête et ses membres sont ossifiés. Je vous épargnerai donc le détail de l'intervention. Sachez que cette opération est souvent insoutenable pour nombre de professionnels. Dans ce contexte, le risque est réel de voir le nombre de médecins volontaires pour réaliser cet acte diminuer, les gestes étant difficiles et dangereux. Nous nous trouverions ainsi dans une situation paradoxale. Alors que l'idée est d'apporter une réponse à un problème réel, le risque serait grand que l'allongement des délais, qui nécessiterait un nombre de praticiens accru, entraîne des délais supplémentaires en raison du refus de médecins de pratiquer de tels actes. actes. Quelles que soient les évolutions de la société, l'IVG demeure un acte d'une nature particulière. C'est la raison pour laquelle à la liberté de la femme de disposer de son corps doit répondre la liberté du praticien d'invoquer la clause de conscience. Le maintien de la clause de conscience spécifique se révèle au demeurant un moyen de protection des femmes, puisqu'en contrepartie le médecin ou la sage-femme concerné doit orienter la patiente vers un confrère. Cette disposition ne pose donc pas de problème, me semble-t-il.

avant de commencer, je souhaiterais remercier Albane Gaillot, à l'origine de cette proposition de loi, ainsi que l'ensemble des députés qui se sont battus pour qu'elle soit adoptée à l'Assemblée nationale. Je souhaite les remercier pour leur travail et pour leur mobilisation sans relâche pour le droit des femmes à disposer de leur corps- puisque c'est au fond de cela, et uniquement de cela, qu'il est question aujourd'hui, comme à chaque fois qu'il est et qu'il sera question d'avortement. Nous avons beaucoup entendu pendant les débats qu'un avortement à quatorze semaines serait plus traumatisant qu'un avortement à douze semaines. Excusez-moi, mais qui évalue cela ? Vous ? Vous ? Vous pensez pouvoir savoir à la place d'une personne enceinte de douze semaines qu'il est plus traumatisant de mettre fin à cette grossesse qu'elle ne souhaite pas poursuivre que de la mener à terme alors qu'elle ne le veut pas ? Je ne comprends pas comment l'on peut se sentir légitime pour apprécier cela- davantage encore, messieurs, quand on n'aura jamais à prendre cette décision. Vous savez quoi ? Vous pensez qu'avorter à quatorze semaines c'est traumatisant. N'avortez pas à quatorze semaines ! La seule chose, c'est que nous, nous ne vous demandons pas votre avis sur ce qui est traumatisant ou pas pour nous. Merci, mais non, merci ! Nous sommes bien assez grandes pour le décider nous-mêmes. Nous, c'est avec des raisonnements pareils, c'est la logique même de notre liberté à disposer de notre corps, sur laquelle est fondé le droit à l'avortement, que vous remettez en cause. Si la boussole, c'est ce que vous, vous pensez de l'impact d'un avortement, comment fait-on ? Il y a des avortements à quinze semaines

Non seulement vous avez une opinion sur ce qui va être le plus traumatisant pour les personnes concernées, mais en plus vous pensez vraiment pouvoir décider qu'un avortement n'aura pas lieu. Vous croyez vraiment que vous avez le pouvoir d'empêcher des personnes d'avoir recours à des avortements quand elles le souhaitent. Je vais vous dire une chose. Cela va peut-être vous décevoir, mais vous n'avez pas ce pouvoir. De la même manière que, lorsque les avortements sont interdits, il y a non pas moins d'avortements, mais plus d'avortements illégaux, donc dangereux ; quand on interdit l'avortement après douze semaines,

quelques mots à présent sur la clause de conscience spécifique. Je suis désolée, mais l'on ne peut pas mettre au même niveau le droit à l'avortement, qui est un droit fondamental, et le droit des personnels soignants à décider des actes qu'ils et elles pratiquent. Ce n'est pas du même niveau. Quand on a, de par sa fonction, le pouvoir matériel de donner accès à un droit fondamental individuel, ce n'est pas de sa conscience personnelle qu'il s'agit. On exécute la décision d'une personne d'exercer ses droits. La clause de conscience générale suffit donc largement. Certes, personne n'avorte par opportunité, par confort ou par envie. Mais l'avortement n'est jamais un problème. L'avortement est une solution à un problème. Les grossesses non désirées, le mauvais accès à la contraception, le manque d'éducation sexuelle, les viols : ils sont là, les problèmes. Un avortement peut être une épreuve difficile- pas toujours, mais il peut l'être. Ce peut être un choix difficile, mais pas toujours. Très souvent, c'est un choix très facile et très rapide. Nous ne sommes pas là pour en juger. Nous sommes là pour protéger un droit fondamental.

madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement, que nous examinons en deuxième lecture, a connu un parcours tumultueux. Déposée par la députée Albane Gaillot, que je salue, du groupe Écologie Démocratie Solidarité, et plusieurs de ses collègues, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 8 octobre 2020, il a fallu attendre novembre 2021 pour que le groupe La République en Marche l'inscrive à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Enfin, après d'ultimes hésitations, le Gouvernement s'est résolu à l'inscrire en deuxième lecture à l'ordre du jour du Sénat. Quels enseignements pouvons-nous tirer de ce cheminement complexe ? Tout d'abord, sans l'impulsion du mouvement féministe en faveur de l'allongement du délai d'avortement et sans le soutien de femmes politiques, ce texte n'aurait jamais été jusqu'ici. À ce titre, je rappelle que le groupe communiste républicain citoyen et écologiste avait déposé en 2017 une proposition de loi visant à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, et qu'en 2019 il en avait déposé une autre concernant notamment l'allongement à quatorze semaines du délai d'accès à l'IVG et la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer des IVG instrumentales. Que de temps perdu pour les femmes ! Le droit à l'interruption volontaire de grossesse est un acquis chèrement conquis, qui, en France comme dans le monde, demeure fragile, et peut être remis en cause à tout moment.

ou encore hier à l'occasion de l'élection à la présidence du Parlement européen de Roberta Metsola, militante déclarée contre l'interruption volontaire de grossesse. Une véritable honte Comment s'étonner, dès lors, de l'opposition de la droite sénatoriale, qui a rejeté la semaine dernière en commission le texte visant l'allongement de l'IVG en utilisant des arguments choquants, d'un autre âge, sans parler de la motion tendant à opposer la question

passant ainsi de douze à quatorze semaines de grossesse ». L'exemple vient d'en haut, l'opposition du Président de la République Emmanuel Macron, qui a récemment rappelé au Pape son opposition personnelle à l'allongement des délais d'interruption volontaire de grossesse. Il est regrettable qu'en 2022, près de cinquante ans après la loi Veil, l'amélioration de la prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse puisse encore déclencher une telle hostilité, de La République en Marche aux Républicains. En attendant, les femmes subissent de fortes disparités territoriales dans l'accès à l'IVG, liées en particulier à la diminution du nombre d'établissements de santé la pratiquant- de 22 % en quinze ans -ainsi qu'à leurs capacités réduites, sans oublier la pénurie de personnel. Le rapport de la délégation aux droits des femmes et

Il faut bien avoir conscience de la diversité des situations des femmes qui dépassent le délai légal pour avoir recours à l'avortement. Malheureusement, mon intervention, bien trop courte, ne me donne pas la possibilité de les aborder. Je remercie le docteur Ghada Hatem-Gantzer, médecin-cheffe de la Maison des femmes de Saint-Denis, pour le travail qu'elle réalise

pour avoir recours à ce droit. On estime leur nombre entre 3 000 et 5 000 chaque année. Enfin, l'allongement du délai d'accès à l'IVG doit s'accompagner de moyens financiers et humains pour les structures réalisant des IVG. Il faudra sans doute aller encore plus loin en matière d'allongement du délai, à l'instar d'autres pays européens.

soyons clairs : il n'est pas question d'opposer deux camps dans cette discussion. L'avortement est un droit fondamental, et aucun d'entre nous n'a envie de le remettre en question. La volonté d'allonger le délai pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse met en lumière deux types de réalités. Les premières sont des inégalités sociales,

L'allongement du délai d'intervention n'est pas le fond du problème : il est urgent dans ce pays de se donner des moyens d'accueillir

qui est actuellement de douze semaines, et que cet acte est considéré par les professionnels de santé eux-mêmes comme d'autant moins anodin qu'il est pratiqué tardivement au cours de la grossesse Considérant que l'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 autorise les sages-femmes, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, à réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissement de santé, et qu'il paraît donc prématuré de pérenniser dès aujourd'hui l'extension de cette compétence aux sages-femmes ; Considérant que le texte transmis au Sénat en seconde lecture renonce à supprimer la clause de conscience spécifique à l'IVG, clause qui figure dans notre droit depuis la loi Veil de 1975 et confirme ainsi le fait que cet acte mérite une considération particulière Considérant que la clarté des débats aurait sans doute gagné, madame la ministre, à ce que le Gouvernement précise sa position sur ce texte avant de prendre l'initiative de l'inscrire à l'ordre du jour du Sénat en deuxième lecture Considérant que le Sénat a déjà rejeté ce texte en première lecture en commission puis, par l'adoption d'une motion tendant à opposer la question préalable, en séance publique ; La commission estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette proposition de loi. La parole

concernées des femmes jeunes, précaires, victimes de violences et éloignées des centres de soins : ces femmes sont les plus susceptibles de ne pas parvenir à interrompre dans les délais légaux une grossesse qu'elles ne souhaitent pas poursuivre.

de pratiquer les IVG médicamenteuses et instrumentales va dans le bon sens, tout comme la téléconsultation. La prise en charge par la sécurité sociale de la contraception féminine jusqu'à 25 ans constitue également

toutefois qu'il « ne saurait cautionner une mesure prise pour pallier les multiples dysfonctionnements matériels, économiques, juridiques d'une politique de santé publique majeure pour les femmes. » Le dépassement du délai légal pour une IVG peut être la conséquence du diagnostic tardif d'une grossesse,

Parce que les nombreux professionnels que j'ai interrogés sont très partagés sur cet allongement. Parce qu'avant d'allonger les délais, on doit garantir l'accès à l'IVG pour toutes les femmes.

de cette utilisation de notre règlement pour faire échec à l'extension des droits des femmes. Le débat aurait pu et aurait dû avoir lieu. Pour toutes ces raisons, et parce que nous soutenons cet allongement du délai, le groupe CRCE votera contre cette motion.

vote. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce matin Emmanuel Macron, Président de la République et président du Conseil de l'Union européenne, tenait un discours devant les eurodéputés. À cette occasion, il a annoncé vouloir inscrire le droit à l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux

cela commence à faire beaucoup. J'aurais pour ma part voté ce texte, et je voterai contre la motion. En effet, des milliers de femmes en France se retrouvent chaque année hors délai et partent pour cette raison avorter à l'étranger.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à démocratiser le sport en France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

dans laquelle je proposais de consacrer sur le plan législatif la plateforme de lutte contre ces manipulations et de déterminer ses modalités d'action, notamment lorsque la manipulation se déroulait dans un contexte international. Je me réjouis donc aujourd'hui de constater que cette consécration législative est devenue une réalité pour permettre à la plateforme de mieux fonctionner, au niveau national comme au niveau international, et pour que notre pays puisse conserver l'avance qu'il avait prise dans la lutte contre la manipulation des compétitions. Au niveau national, la convention signée en janvier 2016 par l'ensemble des membres de cette plateforme s'avérait impuissante à lever un obstacle juridique qui en a empêché le fonctionnement efficace, ne permettant pas à ses membres d'échanger des informations entre eux. Seuls les échanges entre l'Autorité nationale des jeux (ANJ) et le Service central des courses et jeux (SCCJ) étaient autorisés par la loi. C'est donc une excellente chose que de voter cet article aujourd'hui.

La France occupait la vice-présidence du groupe de rédaction et le secrétaire d'État chargé des sports de l'époque, Thierry Braillard, l'avait signée en septembre 2014. Madame la ministre, où en sommes-nous aujourd'hui dans ce processus de ratification ? En tant que présidente du Conseil de l'Union européenne pour le sport, allez-vous remettre le sujet de la ratification par l'Union européenne à l'ordre du jour ? Je

L'objectif est de laisser le soin à chacune des disciplines sportives, par un accord collectif, de définir les modalités de mise en oeuvre de ces contrats de plus longue durée. Un décret devra préciser les conditions d'application propres à la discipline concernant, en particulier, la mention des thématiques qui doivent être abordées par discipline concernant, par exemple, les minima de salaires spécifiques, l'âge maximal de fin de premier contrat professionnel et la continuité de la formation pédagogique, ainsi que les conditions de renouvellement et de prolongation. La parole

cinq ans afin de sécuriser les clubs formateurs, car les centres de formation français sont excellents. Ils le sont tant que les jeunes espoirs fuient à l'issue du contrat de trois ans vers d'autres horizons, attirés par des propositions alléchantes, des contrats longs et d'excellentes rémunérations amendement a donc pour objet de sécuriser les politiques des clubs tout en prévoyant l'encadrement de contrats prolongés par la négociation collective. J'insiste grandement sur la notion d'accord collectif et de dialogue social entre les parties concernées. Je ne peux donc que cautionner le sous-amendement de notre rapporteur rapporteur puisqu'il vise à encadrer le décret qui, lui-même, encadrera les négociations collectives. Elles devront ainsi porter sur un certain nombre de sujets, notamment les minima de salaires spécifiques et leur évolution possible pendant la période du contrat prolongé.

complémentaire du délit de manipulation des compétitions sportives, prévu par l'article 9 du projet de loi. À nos yeux, il s'agit d'une sorte de manque en ce qui concerne le droit du sport.

Cet amendement vise à faciliter la lutte contre les sites illégaux en raccourcissant notamment les délais

en permettant en particulier au président de l'ANJ de dresser, sous le contrôle du juge administratif, une liste noire de sites que les fournisseurs d'accès à internet devront bloquer immédiatement. Cette procédure s'inspire

Elle crée également une obligation renforcée de diffusion pour les grandes compétitions internationales organisées sur le territoire national. Elle vise, enfin, à mettre en place des garde-fous, afin d'éviter que certaines plateformes ne s'approprient le droit à diffuser des événements sportifs d'importance majeure.

la diffusion en accès libre des grandes compétitions internationales, ainsi que des manifestations sportives lors des compétitions internationales auxquelles prend part une équipe ou un athlète français. Je ne développerai pas la longue liste des compétitions

dans les cinq sports les plus diffusés, il fallait, en 2020-2021, payer plus d'une centaine d'euros ! Il est évident qu'il est alors difficile pour bon nombre de personnes- je pense en particulier aux jeunes

qui avaient vocation à lutter contre le piratage. Il nous semble que la lutte contre ce dernier sera d'autant plus efficace qu'un plus grand nombre de manifestations sportives seront en accès libre.

paraît tout à fait pertinente pour préserver la diffusion des retransmissions sportives en clair à la télévision et mieux mettre en valeur, comme il l'a indiqué, les compétitions féminines, mais aussi des événements exceptionnels comme les jeux Olympiques et Paralympiques.

sujet est extrêmement important si nous voulons populariser la pratique sportive féminine. S'il faut saluer l'augmentation importante de la diffusion des épreuves engageant des équipes et athlètes féminines entre 2012 et 2016, supérieur de l'audiovisuel (CSA) avec l'opération « Sport féminin toujours », ces dernières ne représentent encore que 20 % des rediffusions sportives. Comme le soulignait le rapport d'Annick Billon, Céline Boulay-Espéronnier, Victoire Jasmin et Christine Prunaud, la mise en valeur et la médiatisation des sportifs de haut niveau et professionnels

médiatisation permettrait de créer des vocations et encouragerait les jeunes filles et femmes à prendre des licences. Ensuite, elle obligerait les fédérations et les clubs à lever les freins constatés à la pratique, notamment en matière de lutte contre les stéréotypes,

connaîtra le même sort que le précédent ! Nous assistons ces dernières années à la disparition du sport à la télévision en clair. Premièrement, l'obtention des droits sur les jeux Olympiques et Paralympiques par le groupe Discovery a participé

pu profiter de 3 000 heures de diffusion en clair. À l'heure actuelle, le seul engagement pris concerne les heures fixées par le Comité il ne faut pas oublier que le service public audiovisuel a connu un nouveau plan de rigueur. Outre les dégrèvements de redevance estimés à 624 millions d'euros, ce sont près de 200 millions d'euros de crédits qui ont disparu sur le quinquennat, dont France Télévisions a assumé la plus grosse charge. Dans ces conditions, il apparaît difficile pour le groupe, qui augmente par ailleurs ses engagements en matière de production, d'aller se battre contre les chaînes cryptées pour des droits dont le marché constitue une bulle spéculative importante. Troisièmement, nous avons vu arriver de nouveaux opérateurs extrêmement puissants. Si la tentative d'Orange, au début des années 2000, a été un échec, BeIN Sports a montré une décennie plus tard qu'il existait bien un marché. un marché. Après le fiasco Mediapro-Téléfoot, l'arrivée d'Amazon dans le football et les rumeurs autour d'un intérêt de Facebook pour la diffusion sportive laissent craindre un nouveau coup porté à la chaîne cryptée

et j'en profite pour interpeller de manière sportive et amicale notre collègue, M. Bacchi. Compte tenu de son origine géographique, j'ai la faiblesse de penser qu'il est un supporter de l'Olympique de Marseille. S'il veut que, demain, la Ligue des champions revienne au stade Vélodrome,

comprennent les évolutions suivantes par rapport à la rédaction initiale. Premièrement, les décisions de la société commerciale ne pourront être contraires à la délégation

en capital effectués à son profit, soient répartis entre cette société, la fédération sportive délégataire, c'est-à-dire le sport amateur, la ligue et les sociétés sportives. Il faut que la fédération puisse continuer à percevoir

c'est une vision à court terme. J'espère que la ligue, aujourd'hui, travaille sur un projet à moyen et long terme.

Rupert Murdoch l'avait bien compris avec le championnat anglais, et ce dernier est grâce à lui aujourd'hui le premier d'Europe et du monde, et de très loin. Si l'on veut vraiment

explication de vote. Monsieur le rapporteur, j'ai bien noté les efforts de la commission pour essayer d'encadrer quelque peu cette société commerciale, même si

Nous devons encadrer également le management de gestion de la société qui gère les fonds de la société commerciale. Ces précautions sont indispensables si nous voulons que l'intérêt des investisseurs ne repose pas uniquement Il est également souhaitable que la manne financière apportée par cette exploitation entraîne des retombées sur toute la filière, notamment sur le sport amateur et le sport scolaire, qui devrait être le premier vivier de recrutement des futurs joueurs professionnels. Pour faire rentrer l'argent rapidement, les ligues donnent les clés de la maison à l'investisseur, au risque de ne plus avoir la main sur les droits.

est inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée à la suite de cette proposition de loi. Au regard du nombre d'amendements restant sur le texte en discussion et en accord avec la commission des lois et le Gouvernement, je vous propose de prévoir d'ores et déjà de reporter l'examen de la proposition de loi visant à améliorer la à demain, jeudi 20 janvier, à l'issue des conclusions des commissions mixtes paritaires sur le projet de loi relatif à la protection des enfants et sur la proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Il n'y a pas d'observation ?